d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie hier, mercredi 7 novembre, sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

L'ordre du jour appelle l'examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques

à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires,

La procédure accélérée a été engagée sur ces textes. Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Jean-Claude Requier, auteur de la proposition de loi.

le groupe du RDSE a pris l'initiative de soumettre au vote de la Haute Assemblée cette proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Cette agence, je vous le rappelle,

Le chef de l'État avait alors clairement exprimé sa volonté de voir aboutir la création de cette agence, afin de mettre au service des projets des territoires un État facilitateur clairement identifié dans chaque département, avec un interlocuteur unique et la capacité de mobiliser des compétences en ingénierie territoriale. Ce texte est le résultat d'un travail en partenariat entre le groupe du RDSE et le ministère de la cohésion des territoires, alors dirigé par notre collègue Jacques Mézard,

un texte équilibré, prévoyant une synergie organisée avec plusieurs agences : il est en effet chaque jour plus évident que la coordination des diverses politiques de ces dernières est une impérieuse nécessité pour mieux répondre aux légitimes aspirations du territoire, en particulier dans les zones fragiles. Il est plusieurs points que le groupe du RDSE considère depuis l'origine comme fondamentaux. Les modifier serait contraire à l'essence même du travail qu'il a effectué. Tout d'abord, nous avons expressément soutenu, en accord avec l'ancien ministre, que l'agence soit présidée par un élu.

Au moment où le combat contre la fracture numérique est légitimement une priorité nationale pour lutter contre les déséquilibres territoriaux- je salue notamment le travail de Patrick Chaize Patrick Chaize -, il serait anormal que l'Agence du numérique ne rejoigne pas l'ANCT. C'est d'ailleurs une orientation énoncée par le Président de la République lui-même. Nous connaissons les réticences celles de Bercy et d'autres clairement identifiées qui, de manière directe ou indirecte, empêchent cette fusion ou à tout le moins la retardent, pour chercher à y échapper. Aucun des arguments exposés ne repose sur des fondements solides. L'enjeu est pourtant clair : veut-on ou non que le développement du numérique sur l'ensemble du territoire soit une ambition partagée entre les collectivités locales et l'État pour un aménagement équilibré du territoire,

Je sais que M. le rapporteur, Louis-Jean de Nicolaÿ, dont je salue de travail considérable, partage lui aussi cette préoccupation majeure. Bien sûr, nous attendons une confirmation claire du Gouvernement sur ce point et nous espérons qu'il maintiendra la même position devant l'Assemblée nationale. Plus globalement, l'administration territoriale de l'État a été confrontée ces dernières années à des transformations géographiques et démographiques profondes, notamment en raison du poids plus prépondérant des métropoles. les collectivités territoriales ont dû digérer cette évolution, mais aussi faire face à des transferts successifs de compétences, sans pour autant bénéficier des compensations financières correspondantes, ce qui a pénalisé les plus fragiles

l'ATESAT, a ainsi été, à notre sens, une erreur. Dans son rapport public thématique sur les services déconcentrés de l'État, la Cour des comptes estime que le bilan global de cette suppression pourrait être défavorable en termes d'efficience comme d'impact sur l'ensemble des finances publiques. Les Les collectivités territoriales, du moins celles qui le peuvent, ont été obligées de compenser la perte de ces moyens d'ingénierie publique. Mes chers collègues, notre pays doit franchir une nouvelle étape dans le renforcement de la légitimité de l'action publique pour rétablir une relation de confiance avec nos concitoyens. L'État doit faciliter et accompagner les projets en partant des besoins des territoires. Telle que nous la concevons, la présence de l'État dans nos territoires ne doit pas se diluer dans un maquis normatif souvent incompris. L'État ne doit pas être celui qui répond sans apporter de solutions. Au contraire, Au contraire, il doit soutenir la libre autonomie des collectivités territoriales, leur développement économique et l'accessibilité des services publics, en proposant des solutions. Pour cela, l'action publique doit se moderniser. Des changements culturels s'imposent, dans une logique de guichet unique très clairement détaillée dans le rapport Morvan. L'ANCT doit être un instrument de mise en cohérence opérationnelle des moyens techniques, juridiques, financiers et humains, assurée par le préfet. À la fois délégué territorial de l'agence et représentant de l'État, celui-ci disposera d'une vision d'ensemble sur l'appui qui pourra être apporté aux territoires, surtout à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour nous une verticalité inversée que je qualifierais de vertueuse. Nous n'avons surtout pas la volonté de mettre en oeuvre une recentralisation de la décision : cela n'irait pas dans le sens de l'histoire. Il est d'ailleurs intéressant de s'arrêter sur la définition d'une agence telle qu'elle a été posée par le rapport du Conseil d'État publié en 2012 l'agence est un organisme autonome exerçant une responsabilité structurante dans la mise en oeuvre d'une politique nationale. À ce titre, elle concourt à la mise en oeuvre de la politique de la Nation au sens de l'article 20 de la Constitution. Cet excellent rapport prévoyait quatre critères pour un recours approprié aux agences. Nous les avons appliqués : l'efficience, avec une spécialité dans des tâches de gestion à grande échelle ; l'expertise, distincte de celle des services de l'État et que nous avons mobilisée dans sa diversité, à l'instar de ce que préconisait le rapport Morvan ; le partenariat avec les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire ; et, enfin, la neutralité en évitant l'intervention du pouvoir politique dans l'ensemble des processus de décision. Le recours à une agence se justifie donc pour permettre à l'État de se concentrer sur son rôle de stratège. Comme l'écrivait Alexandre-François Vivien en 1845 dans un ouvrage consacré à la science administrative

La gouvernance laisse ainsi une place prépondérante aux représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels sera élu le président du conseil d'administration. Nous étions d'ailleurs très défavorables à la mise en place d'un duo entre le directoire et le conseil de surveillance, qui aurait, selon nous, réduit les pouvoirs des représentants des collectivités territoriales. L'ANCT ne devra certainement pas être une énième structure administrative ni une coquille vide. Elle devra mutualiser des moyens pour surmonter l'organisation aujourd'hui en silo qui pénalise la conduite des projets. Comme le souligne à juste titre le Conseil d'État dans son avis dont nous avons voulu la publication, il reviendra ensuite au pouvoir réglementaire de définir « des procédures de décision efficaces permettant au nouvel organisme de répondre aux attentes des collectivités territoriales et d'assurer pleinement sa mission de coordination des actions et projets des autres services et opérateurs de l'État. Dans tous les cas, le Conseil d'État a jugé positive cette orientation opérationnelle. Pour conclure, je salue le travail du rapporteur et de la commission, grâce auquel a été apporté un certain nombre d'améliorations à la suite de l'avis du Conseil d'État. Toutefois, nous exprimerons dans le cours de la discussion une opposition au report à 2021 de la date d'intégration de l'Agence du numérique. Nous le savons : ou bien elle est intégrée dès le départ ou bien cette intégration ne se fera pas. C'est d'autant plus vrai si cette intégration doit intervenir un an avant l'échéance du plan France très haut débit. Mes chers collègues, Mes chers collègues, cette agence est très attendue par les collectivités territoriales, en particulier par les plus fragiles d'entre elles. Le Sénat est aujourd'hui dans son rôle de représentant des collectivités territoriales. Honorons ce mandat qui nous a été confié en faisant de cette agence un outil efficace d'aménagement du territoire et un instrument à l'écoute de chaque territoire

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis l'annonce de la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires par le Président de la République en juillet 2017, lors de la Conférence nationale des territoires, une longue période s'est écoulée. Il a fallu en effet attendre près d'un an après cette annonce pour que le Premier ministre confie au préfet Serge Morvan, que je salue, la mission de rédiger un rapport de préfiguration de cette agence. Ce rapport, remis en juin dernier, a été rendu public tardivement et de manière curieuse puisque nous en avons pris connaissance une publication sur un site internet par une organisation syndicale. dit projet de loi ÉLAN, il y a quelques semaines, le Gouvernement a déposé au dernier moment un amendement visant à autoriser la création de cette agence par voie d'ordonnance. Le Sénat, trouvant cette procédure quelque peu cavalière, a rejeté cet amendement. Début octobre, nous avons constaté l'inscription à l'ordre du jour, en procédure accélérée, d'une proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires déposée par notre collègue Jean-Claude Requier J'ai donc souhaité avec Jean-Claude Requier déposer une proposition de loi organique visant à prévoir l'audition, en application de l'article 13 de la Constitution, du directeur général de l'agence par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il nous a paru effectivement indispensable, dès lors que cette agence serait créée, de prévoir un avis du Parlement sur la nomination de son directeur général, comme c'est le cas pour la plupart des organismes comparables. Le dépôt de cette proposition de loi organique ne constitue donc en rien un blanc-seing pour la création de l'agence nationale telle qu'elle est prévue par la proposition de loi initiale. J'ai en effet eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises, depuis l'annonce de la création de cette agence, qu'une telle structure n'aurait de sens et d'intérêt que dans la mesure où elle serait réellement utile aux collectivités locales et aux territoires, ce dont je ne suis hélas pas convaincu L'essentiel pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'est pas de créer un outil, quand bien même il serait pertinent. L'essentiel, pour nous, est que l'aménagement du territoire cesse enfin d'être le parent pauvre des politiques publiques et qu'il y ait une véritable volonté en termes d'aménagement du territoire.

sur le manque de volonté politique en matière d'aménagement du territoire et sur le creusement des fractures territoriale et sociale qui en découlent. Nous avons présenté ce rapport à Jacques Mézard, votre prédécesseur, madame la ministre. Nous en avons débattu ici même le 25 octobre 2017 nous vous avons également remis en main propre ce document la semaine dernière en commission. Nous espérons que vous en ferez le meilleur usage possible, mais jusqu'à présent force est hélas de constater que nos travaux ont peu inspiré l'action du Gouvernement Madame la ministre, vous avez, lors de votre audition devant la commission, prôné le parler-vrai. Mais où est le parler-vrai quand le Président de la République et le Gouvernement disent vouloir renouer avec les territoires et les élus locaux alors que les crédits de la cohésion des territoires n'augmentent que pour la politique de la ville ? Vous le savez, madame la ministre, les déclarations d'amour ne suffisent pas : il faut des preuves d'amour. Or, pour l'instant, nous ne les voyons pas encore

Au-delà de ces constats, j'insisterai sur trois points. Première remarque, le Gouvernement doit prendre ses responsabilités concernant la création de cette agence et ne doit pas se cacher derrière une proposition de loi. de loi. Je m'étonne que l'ambition affichée par le texte qui nous est soumis avec le soutien de l'exécutif soit très en deçà des ambitions exprimées par le préfet Morvan dans son rapport de préfiguration réalisé à la demande du Premier ministre. Premier ministre. Pourquoi un périmètre si réduit a-t-il été choisi ? Pourquoi un tel manque d'ambition ? Dans ces conditions, quels sont l'intérêt et l'utilité de cette agence ?

! Nous sommes nombreux à demander la mise en place d'un guichet unique pour les collectivités territoriales, mais il convient également de simplifier fortement les contraintes pesant sur les porteurs de projets locaux.

La question des ressources dont bénéficiera l'agence est également essentielle. Sur ce point aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. L'agence fonctionnera-t-elle à moyens constants ou avec des moyens supplémentaires ? Le Gouvernement envisage-t-il de joindre la parole aux actes et de débloquer des financements pour soutenir les territoires au travers de cette agence ? J'ai cru comprendre en vous écoutant, madame la ministre, lors de votre audition que nous devrions attendre le projet de loi de finances pour 2020

Je vous invite à la plus grande prudence, car la DETR est une dotation fondamentale pour la cohésion des territoires. Il ne faudrait pas déshabiller la DETR pour habiller l'agence nationale de la cohésion des territoires. Deuxième remarque, si je me félicite que le numérique soit désormais reconnu comme un élément essentiel de la cohésion des territoires- au point que l'Agence du numérique est l'une des rares structures à intégrer partiellement cette nouvelle agence -, ce n'est pas le plus important et surtout ce n'est pas suffisant.

que la question serait réglée dans les deux à trois ans, et la réalité, il y a non pas un fossé, mais un gouffre ! Madame la ministre, si le Gouvernement ne change pas de braquet et continue uniquement à se glorifier d'un accord prétendument historique avec les opérateurs, à la fin de ce quinquennat, on sera très loin d'une réelle couverture en téléphonie mobile, comme nous l'annonce sans cesse le Gouvernement. Par manque de temps, je n'évoquerai pas le très haut débit fixe et les craintes qui pèsent sur son financement. Là encore, la fermeture du guichet qui était destiné à financer le déploiement de la fibre est source plutôt d'inquiétude que d'espoir. Enfin, ma troisième remarque vise à souligner le travail effectué sur ce texte par la commission que j'ai l'honneur de présider, tout particulièrement par le rapporteur, Louis-Jean de Nicolaÿ,

de l'agence ; améliorer la prise en compte des territoires les plus fragiles, qui sont ceux qui ont aussi le plus besoin de cette agence. La commission souhaite que cette agence apporte une véritable plus-value aux territoires, mais les incertitudes sur son périmètre et sur ses moyens sont encore nombreuses.

à M. le rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet d'agence nationale de la cohésion des territoires prévu par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'est pas nouveau

Le Président de la République avait saisi la balle au bond- si je puis m'exprimer ainsi -et annoncé la création prochaine d'une telle structure, d'abord lors de la Conférence nationale des territoires, qui s'est tenue au Sénat le 17 juillet 2017, puis devant le Congrès des maires de France, le 24 novembre 2017. L'annonce L'annonce a ensuite été confirmée à plusieurs reprises par le Gouvernement, que ce soit par la voix de Jacques Mézard, de Julien Denormandie ou par vous-même, madame la ministre. Alors que nous nous apprêtons à examiner le contenu de la proposition de loi, je souhaite vous faire part de trois remarques liminaires. sur la méthode, que je regrette. Les atermoiements du Gouvernement ont conduit légitimement certains de mes collègues à anticiper sur les projets gouvernementaux. Je pense, par exemple, à la proposition de loi déposée en octobre 2017 à l'Assemblée nationale par notre collègue Philippe Vigier et, bien sûr, à la proposition de nos collègues Philippe Bas, Bruno Retailleau et Mathieu Darnaud, adoptée par le Sénat le 13 juin dernier. Plus récemment, il y a eu une tentative du Gouvernement de se voir habiliter à légiférer par ordonnance pour créer l'agence, à l'occasion de l'examen du projet du projet de loi ÉLAN en séance au Sénat. Cette initiative intervenait alors même que le préfet Serge Morvan, ancien directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et cinquième commissaire général à l'égalité des territoires en quatre ans, avait été chargé quelques semaines plus tôt par le Premier ministre de préfigurer la création de cette agence. Au-delà de l'absence d'étude d'impact, puisque nous examinons aujourd'hui une proposition de loi, la concertation aurait dû être plus importante. J'ai eu à peine quatre semaines pour travailler sur ce texte, consulter une douzaine d'organismes et préparer les vingt-trois amendements que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adoptés lors de sa réunion du mercredi 31 octobre dernier. Dans ce contexte, il est heureux que le président du Sénat ait recouru à la faculté que lui offre le dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution de saisir le Conseil d'État, afin que ce dernier rende un avis sur les dispositions de la présente proposition de loi. Cet avis a utilement éclairé mes travaux. En outre, les échanges que j'ai eus avec Alain Lambert, président du Conseil national d'évaluation des normes, ont révélé l'impréparation du Gouvernement quant à la simplification des procédures imposées aux collectivités. Deuxième remarque, si l'expérience de l'agence nationale de la cohésion des territoires s'avère concluante, cette structure pourrait permettre une véritable rationalisation des actions de l'État dans les territoires avec, à la clé, évidemment, nous l'espérons, une économie pour les finances publiques. Mais l'ambition du texte qui nous est soumis et celle du Gouvernement semblent en deçà des attentes de nos concitoyens et des élus locaux. Les fractures françaises sont nombreuses et bien connues dans l'accès au numérique, dans l'accès aux soins, avec la problématique des déserts médicaux, dans l'accès aux services publics et dans le domaine de la mobilité, mot cher à notre collègue Mathieu Darnaud. Autant de freins à la cohésion et à l'ascension sociales Je me réjouis, à cet égard, de l'examen prochain du projet de loi d'orientation des mobilités par notre assemblée, car les mobilités sont autant de leviers pour soutenir les territoires les plus fragiles. Je ferme cette parenthèse en regrettant que le Gouvernement n'ait pas décidé, en amont, d'adopter une approche décloisonnée concernant les missions de l'agence, concept dont nous entendons souvent parler ces derniers temps, mais qui peine à se matérialiser. troisième remarque. L'État doit prendre ses responsabilités sur un certain nombre de volets. Je pense, en particulier, à la question des ressources dont bénéficiera l'agence, au sujet de laquelle la frilosité du Gouvernement conduit à s'interroger, mais aussi à la question de l'association des élus locaux et nationaux à sa gouvernance. En clair, les territoires doivent être considérés par l'État comme des partenaires égaux. À ce titre, j'attire l'attention du Gouvernement sur le fait que le financement de l'agence ne devrait en aucun cas venir en soustraction des moyens actuellement accordés aux collectivités territoriales.

Il est inenvisageable que le Gouvernement revienne sur les engagements pris concernant la ressource DETR. Ce que les territoires attendent, ce sont des moyens supplémentaires pour les accompagner, et non des tours de passe-passe à périmètre budgétaire constant. Lorsque l'on donne d'une main et que l'on reprend de l'autre, cela finit toujours par se voir. Les élus ne sont pas dupes, vous en savez quelque chose ! Ces remarques formulées, je souhaite vous présenter la logique du texte adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui s'organise autour de quatre objectifs principaux. Premièrement, la commission a souhaité renforcer le rôle des élus locaux et nationaux, en améliorant la gouvernance nationale et locale de l'agence. La composition du conseil d'administration a été revue et un comité local de la cohésion territoriale institué. Deuxièmement, la commission a souligné la nécessité, pour l'agence, de s'intéresser aux territoires les plus en difficulté. L'agence ne doit pas s'adresser aux grandes métropoles disposant de capacités techniques importantes. Elle doit servir en priorité les territoires ruraux et périurbains, qui souffrent d'un abandon reconnu. Troisièmement, la commission a souhaité assurer dans les meilleures conditions l'intégration de l'Agence du numérique, en sécurisant la période de transition. Sur ce sujet, qui a suscité de nombreuses inquiétudes, dans des délais très contraints, la commission a proposé une première solution, qui pourra encore faire l'objet d'ajustements quand nous l'aborderons, à l'article 2. Au-delà, la commission a également ouvert la voie à un regroupement futur d'autres établissements publics au sein de l'agence. S'agissant des questions de structure, gardons-nous des postures et ayons en tête l'intérêt, pour les territoires, de s'adresser à un interlocuteur unique, dans un souci de bonne utilisation des deniers publics et d'efficacité de l'action publique. Enfin, sans dénaturer le travail effectué par notre collègue Jean-Claude Requier, que je salue, la commission a souhaité procéder à la codification des dispositions relatives à l'agence au sein du code général des collectivités territoriales, pour des motifs de clarté et d'intelligibilité du droit. veux apporter une précision sur le rôle de l'agence : l'ANCT ne sera pas un passage obligé pour les collectivités, pour ne pas affaiblir leur autonomie. Il s'agit d'un outil à la disposition des territoires. Son succès dépendra de l'efficacité de son action, de la rapidité de traitement des dossiers portés par les collectivités territoriales et de l'association des élus et des citoyens à ses interventions. Le déploiement de la fibre optique, l'amélioration de la couverture mobile, la restructuration commerciale et artisanale de nos bourgs, la transition écologique, le renforcement territorial de l'accès aux soins sont aujourd'hui au coeur des préoccupations de nos concitoyens, tout comme la rénovation de l'habitat.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le rapporteur, monsieur l'auteur de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, trois semaines après ma prise de fonctions au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je suis particulièrement heureuse d'être présente devant la Haute Assemblée pour examiner la proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, déposée par le groupe du RDSE. Je tiens dès à présent à saluer le président de ce groupe, le sénateur Jean-Claude Requier, pour cette initiative naturellement bienvenue.

disposant que le directeur général de l'ANCT est nommé par décret après avis des commissions parlementaires compétentes, ce à quoi le Gouvernement ne peut être que favorable. La proposition de loi portant création de l'ANCT est un texte essentiel pour les territoires, leurs élus et, bien sûr, pour l'État.

à une demande formulée par les représentants d'élus, en particulier par François Baroin, président de l'Association

des craintes ou des erreurs de compréhension. C'est pourquoi je tiens dès à présent à dissiper certains malentendus et à vous apporter des précisions sur la méthode, car la création de cette agence traduit avant tout

ils sont confrontés à un certain maquis administratif, qui les contraint à « faire la tournée » de ces opérateurs, qui, nous le savons, interviennent aujourd'hui

C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui, et ce sont les élus de terrain qui le disent, d'un outil de coordination des opérateurs de l'État qui soit, en réalité, un guichet unique- l'expression a été utilisée par M. le rapporteur -vers lequel les élus puissent se tourner pour réaliser leurs projets.

précision : au plan local, c'est le préfet qui sera le délégué territorial de l'agence. Il s'agit là d'un point essentiel, sur lequel je souhaite m'arrêter quelques instants.

territoires. Le préfet sera le représentant unique de l'agence pour les élus locaux porteurs de projets et aura pour mission de fédérer les actions de l'État autour de ces projets. Cela me semble assez simple et me permet de faire le lien avec une autre question récurrente : qui sont ces élus locaux porteurs de projets au profit desquels l'agence interviendra ? Tout simplement

cette politique différenciée, qui tient compte des spécificités de chaque territoire pour assurer son développement, sera au coeur de l'action que je mènerai à la tête de mon ministère.

Alors, oui, je veux que l'État soit en priorité aux côtés des territoires les plus fragiles, pour résorber les fractures territoriales de notre pays. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous vous interrogez également sur la nature de cette aide sur mesure qui sera apportée par l'ANCT. Je tiens là aussi à éclairer un certain nombre de points.

à apporter des capacités techniques pour répondre aux projets des collectivités territoriales et des territoires, surtout de ceux qui ne disposent pas de moyens techniques. Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà des interrogations méthodologiques, auxquelles j'espère avoir répondu, je sais que les enjeux relatifs au périmètre de l'agence, à sa gouvernance, mais aussi aux outils financiers ont fait l'objet de discussions lors de l'examen du texte en commission et ne manqueront pas d'être largement débattus dans cet hémicycle. En la matière, le Gouvernement est favorable à l'équilibre qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi,

et de l'Agence du numérique. L'intégration de ces organismes est un choix pragmatique et stratégique, qui permettra à l'ANCT d'être rapidement opérationnelle

aurait alimenté de longs débats organiques pour fusionner des organismes au statut très divers, ce qui n'aurait pas manqué de compliquer l'action de l'agence. Et, parce que le Gouvernement sait à quel point la couverture numérique du territoire est un élément fondamental de la cohésion et du développement du territoire, il ne peut pas partager la proposition de votre commission consistant à reporter d'une année l'intégration de l'Agence du numérique. C'est pourquoi il défendra un amendement visant à cette intégration dès la création de l'ANCT. En matière de gouvernance, le Gouvernement salue la préservation des équilibres tels que figurant dans le texte initial, à travers un conseil d'administration et un comité d'action territoriale. s'agissant de la création d'une agence de l'État, il ne peut pas être favorable à un partage égal des sièges entre les représentants de l'État et les autres membres du conseil

soient réunies. Au-delà, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements tendant à compléter et à enrichir le texte initial et celui qui est issu des travaux de votre commission. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre eux feront l'objet d'un large consensus.

C'est dans cette optique que l'État se tient aux côtés des collectivités pour faire réussir les projets des territoires. Nous avons identifié, bien sûr, un certain nombre d'« irritants », pour reprendre le terme de mon collègue Sébastien Lecornu, mais, avec l'ANCT, nous avons l'opportunité de créer un nouvel outil lisible et fonctionnel au profit des territoires et des élus

que ceux qui agissent pour et dans les territoires soient plus efficaces et parviennent à réaliser leurs projets. Autrement dit, les fonctionnaires de l'État, dans leur diversité et leurs spécialités, seront mobilisés et fédérés pour aider les projets des collectivités territoriales ou des territoires. Bien évidemment, nous pensons que ce sont les territoires les plus démunis qui seront les plus demandeurs. Je ne doute pas que la richesse du débat qui s'ouvre au sein de votre assemblée

Les deux présidents de ces départements étaient présents, ainsi que le président de la région Hauts-de-France, qui a été le principal interlocuteur de cette négociation avec le préfet de région.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, le présent texte était attendu, et l'histoire mouvementée de sa genèse révèle l'oecuménisme politique de cette attente. Dès 2017, le président de la Haute Assemblée appelait de ses voeux la création d'une agence de la cohésion des territoires, voeux que le Président de la République fit ensuite siens, avant qu'ils ne soient repris par Philippe Vigier et ses collègues députés à l'Assemblée nationale,

C'est là que les choses se corsent quelque peu parce qu'à la lecture du texte qui nous est soumis, la réponse n'est pas des plus évidentes. En effet, ce qu'attendent les collectivités, les collectivités, c'est de pouvoir disposer d'un interlocuteur unique les aidant à mettre en oeuvre leurs projets d'aménagement et de développement territoriaux. Cette attente est particulièrement forte du côté des territoires ruraux, qui réclament à cor et à cri des moyens financiers et humains équitables par rapport aux territoires urbains, la simplification des normes, la possibilité d'expérimenter ; ils demandent aussi que l'on fasse enfin confiance aux élus.

Pourquoi intégrer uniquement les trois premiers établissements et seulement associer les quatre autres ? Par exemple, pourquoi ne pas également intégrer le CEREMA à l'agence ? Un indice : tandis que l'Agence du numérique ne représente que 30 emplois et l'EPARECA 40, le CEREMA emploie près de 3 000 personnes. Il aurait en conséquence été plus compliqué d'intégrer ce dernier à l'agence dès le départ. Le choix du périmètre actuel semble donc purement pragmatique. Il faut se demander : tel établissement, combien de divisions ? Cela, nous pouvons le comprendre. Mais, puisqu'il est décidé de créer l'agence autour du Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, pourquoi faire subsister un petit bout de celui-ci à côté de l'agence ? Pourquoi ne pas le mettre en extinction, comme l'EPARECA ? Est-il pertinent d'intégrer l'Agence du numérique ?

Autrement dit, en l'état actuel du texte, la création de cette agence revient seulement à transférer 40 emplois, ceux de l'EPARECA, dans le CGET. Le texte permettra sans aucun doute une meilleure coordination entre les opérateurs étatiques, ce qui est déjà un progrès. Il y a d'autres raisons de soutenir cette proposition de loi. L'une des principales concerne l'ingénierie. Madame la ministre, vous nous avez expliqué que l'agence servirait à combler les lacunes en ingénierie sur le territoire, ce dont ont vraiment besoin les petites collectivités. De plus, le texte a été amélioré en commission pour intégrer la préoccupation environnementale et pour affirmer que l'aide aux territoires ruraux serait au coeur de l'action de l'agence. Enfin, la proposition de loi organique d'Hervé Maurey garantit que le Parlement conserve un droit de regard sur la gouvernance de l'agence. Même si de nombreuses questions restent en suspens, comme celle de la déclinaison de l'action de l'agence sur le territoire-

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous félicitons que ce sujet soit de nouveau débattu devant notre assemblée. Qui mieux, en effet, que le Sénat pour donner naissance à une agence des territoires Il est de notre devoir constitutionnel de proposer aux élus locaux une institution utile et conforme à leurs attentes. Si cette proposition de loi ne répond pas à tous les espoirs,

En attendant, nous soutenons une coordination renforcée entre la nouvelle agence et l'ADEME, l'ANRU, l'ANAH, la Caisse des dépôts et consignations et les agences régionales de santé, Au-delà des aspects financiers, il y a surtout des problématiques techniques pour concrétiser les projets. L'agence pourra ainsi mobiliser les ressources dont disposent l'État et les opérateurs au profit des porteurs de projets locaux en matière de couverture numérique, de mobilité ou d'environnement. Pour conclure, monsieur le ministre

L'agence pourra ainsi mobiliser les ressources dont disposent l'État et les opérateurs au profit des porteurs de projets locaux en matière de couverture numérique, de mobilité ou d'environnement.

de meilleures relations entre l'État et les collectivités et davantage de ressources pour les élus. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants-République et Territoires soutiendra cette proposition de loi du

lui adresse mes félicitations pour sa nomination à la tête de ce grand ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales-

aux problématiques d'aménagement du territoire. Ce matin et cet après-midi, nous allons discuter d'une proposition de loi qui vise à traduire un engagement présidentiel, à savoir la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires Une agence au service des projets ! Ce texte déposé par M. Jean-Claude Requier et nos collègues du groupe du RDSE porte une double ambition d'une part, faciliter la conception et la réalisation des projets territoriaux envisagés par les équipes municipales, notamment dans les territoires les plus en difficulté ; d'autre part, renforcer les relations entre les services déconcentrés de l'État et les représentants locaux pour une meilleure efficacité. Cette structure, annoncée lors de la Conférence nationale des territoires qui s'est tenue au Sénat en 2017, puis devant le Congrès des maires de France il y a maintenant un an, est, cela a été rappelé, la traduction législative d'une volonté exprimée par les élus. Que sa création soit engagée par une initiative parlementaire, et non par le biais d'un projet de loi, me paraît être, là encore, un signal positif.

Oui, on nous l'a dit, cette agence est désirée, attendue par tous les élus. En premier lieu, par celles et ceux qui sont à la tête des territoires les plus fragiles et/ou les moins richement dotés en moyens financiers et techniques. Nous le voyons d'autant plus clairement aujourd'hui dans le doute, voire le désarroi, d'un certain nombre d'élus- en particulier dans les petites et très petites communes -, qui demandent un accompagnement renforcé pour exercer au mieux leur mandat en portant toujours une ambition forte pour leurs territoires. Mais vous connaissez, autant que nous, monsieur le ministre, mes chers collègues, le climat de méfiance qui peut exister dans nos collectivités territoriales par rapport à ce qui vient de l'État. Cette nouvelle structure, qui en regroupera plusieurs et conventionnera avec d'autres, devra endosser des rôles différents selon les politiques territoriales préexistantes. Là où, par exemple, un département a déjà mis en place des outils d'accompagnement, une question se pose sur le terrain, et je l'entends souvent : comment se fera l'articulation avec l'agence, le préfet délégué de cette dernière et l'exécutif du département, qui s'est déjà beaucoup investi ? Ces clarifications, territoire par territoire, projet après projet, seront nécessaires. Elles seront l'objet, je le crois, de nombreuses prises de parole aujourd'hui.

C'est bien le juste équilibre, le juste dosage, qu'il faudra rechercher. Alors, les élus pourront, en pleine confiance, se tourner vers cette agence. Alors, l'État sera vu non pas comme trop prescriptif, mais bien comme ce qu'il doit être : un accompagnateur et un facilitateur. Alors, l'agence nationale de la cohésion des territoires jouera pleinement son rôle, à savoir combler les manques d'ingénierie et apporter une aide concrète aux élus dans les territoires les plus en difficulté. Je note d'ailleurs un certain nombre d'éléments rassurants à l'article 2. Ainsi, l'agence n'interviendra qu'après accord des conseils municipaux. Elle pourra jouer un rôle essentiel dans les opérations de requalification des centres-bourgs ou dans le déploiement du plan France très haut débit.

Nous serons par la suite vigilants, chacune et chacun dans nos départements, à la mise en oeuvre des actions essentielles à la redynamisation des territoires qui aujourd'hui se sentent déclassés par rapport aux territoires métropolitains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Sur la forme, nous ne pouvons que regretter le passage par une proposition de loi, qui prive les parlementaires d'une indispensable étude d'impact et de l'avis du Conseil d'État. Nous soulignons la réactivité du président du Sénat, qui nous a permis de disposer dans des délais extrêmement courts de cet avis. Pourtant, le fait que le Gouvernement ait déjà déclaré l'urgence sur cette proposition de loi témoigne qu'en réalité, il s'agit bien d'un projet de loi déguisé. Absolument Sur le fond, tout le monde sera d'accord sur le constat alarmant d'une perte d'ingénierie dans les territoires et d'un accroissement des fractures territoriales mettant à mal l'égalité républicaine. L'idée de proposer aux collectivités un nouvel outil est donc plutôt positive. Mais est-ce réellement de cela qu'il s'agit ? Il ne faut pas oublier le contexte. Premièrement, le Gouvernement, qui propose la création de cette agence, poursuit la politique de réduction de l'emploi public, tant au sein des collectivités, par la baisse des dotations, que dans les services de l'État.

Comment faire mieux avec toujours moins ? Nous craignons donc que la création de cette structure ne serve simplement de cache-misère, fonctionnant à coût constant et ouvrant la voie à des mutualisations et à une fongibilité des crédits. Tour de passe-passe utile en période de disette budgétaire ... À ce titre, il faut souligner que le Conseil d'État estime dans son avis « qu'il conviendra que l'agence soit dotée, tant au plan national que local, des ressources suffisantes ». Nous en sommes très loin puisque, de manière incompréhensible, la question des ressources reste en suspens. Or, à défaut d'engagement financier nouveau, cette agence sera simplement une nouvelle couche dans le millefeuille territorial, « machin » de plus qui ne réglera pas les difficultés des territoires en termes de proximité, de maintien des services publics, de présence hospitalière, éducative et judiciaire, de développement d'un réseau de transport ou numérique Quel accès pour les collectivités les plus fragiles et les communes rurales ? Cette agence n'est donc pas la baguette magique du retour de l'État au sein des territoires. Pour cela, il faudrait, loin des politiques gouvernementales actuelles, mener une politique offensive d'investissement public et de soutien réel aux collectivités, soutenir avec une ingénierie dédiée et de proximité les initiatives, l'innovation et le dynamisme de nos territoires. Nous avons également des inquiétudes sur les modalités retenues pour la création de cette agence. Premièrement, nous estimons que son statut devrait être celui d'un établissement public administratif fonctionnant avec des personnels fonctionnaires ou sous contrat public, afin d'affirmer la dimension d'intérêt général des missions de l'agence, à l'opposé d'une vision presque exclusivement commerciale. Nous nous inscrivons ainsi en faux avec la conception, soutenue dans le rapport de Serge Morvan, d'une logique de guichet faisant face à des « clients ». Les mots utilisés en disent long pour ce qui concerne les missions de cette agence, car la proposition ne va pas aussi loin que le rapport Morvan en termes d'intégration des opérateurs de l'État, notamment de l'ANRU et de l'ANAH. Pourtant, nous sommes inquiets. Alors que le CGET est intégré dans cette agence, nous constatons qu'il n'est fait aucune mention de la politique de la ville dans les missions de cette dernière. Pourquoi ce trou noir ? Qui s'occupera demain de ces politiques ? Nous proposerons donc de reprendre très explicitement toutes les missions du CGET, à l'exclusion bien sûr de ce qui relève de l'administration centrale, au sein des compétences de la future agence. Nous sommes d'ailleurs dubitatifs : l'ensemble de la politique de cohésion des territoires serait confié à cette agence. Nous estimons pourtant que l'État conserve une responsabilité première en la matière. L'État ne saurait être seulement un guichet. La puissance publique doit offrir une vision, un cadre et les outils pour atteindre des objectifs, outils définis avec le concours de la représentation nationale. La création de l'agence ne peut donc s'accompagner d'une déresponsabilisation de l'État ou d'une multiplication des partenariats public-privé, comme le permet la possible filialisation de la future agence. Enfin, cette agence se place, non pas dans une volonté de décentralisation, mais dans une vision très verticale du pouvoir. Ce n'est en réalité qu'une déconcentration renforcée autour d'un préfet de département qui devient omnipotent, seul interlocuteur pour les élus locaux. Par ailleurs, cette nouvelle agence, en se plaçant dans la position d'un guichet unique, reste dans cette même logique de collectivités usagères et non coconstructrices de politiques publiques. Nous proposerons, à l'inverse, de rendre majoritaire la représentation des collectivités et des élus locaux dans le conseil d'administration de l'agence, les femmes et les hommes a d'ores et déjà été retenue par le rapporteur, sur notre initiative. Pour retrouver de la sérénité, les rapports entre l'État et les collectivités doivent être fondés sur une confiance renouvelée et renforcée dans les collectivités. Face aux enjeux climatiques, nous sommes tous conscients que la transition écologique et énergétique doit passer par les territoires qui sont les plus proches des citoyens, c'est-à-dire les communes et intercommunalités. Nous estimons qu'il convient d'ouvrir une nouvelle phase de décentralisation, mais avec des moyens financiers, humains et techniques de proximité. Il faut sortir du « tout privé », qui se désintéresse de l'intérêt général et de l'égalité républicaine. Les territoires ne peuvent être jugés sous le seul angle de la compétitivité. Les mots ont leur importance. Or il n'est fait que peu de cas dans ce texte, tout comme dans le rapport Morvan, des habitants, des élus, des associations qui agissent au quotidien pour rendre nos territoires vivants, innovants et vertueux. Le mot « cohésion » a pris la place des mots « égalité » et « équité » pour ce qui est des territoires ; nous le regrettons

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires comme interlocuteur privilégié des collectivités territoriales en matière d'ingénierie répond à une attente forte des territoires fragiles. Aussi, le groupe socialiste et républicain y souscrit pleinement dans son principe. Avant d'en venir au fond, permettez-moi de revenir, à mon tour, sur les conditions de l'examen de cette proposition de loi. Dans son discours du 17 juillet 2017 prononcé au Sénat, le Président de la République avait annoncé la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, confirmée quelques mois plus tard à Cahors par le Premier ministre. Une mission de préfiguration a donc été confiée à M. Serge Morvan, que je salue. Parallèlement, le groupe majoritaire du Sénat avait pris l'initiative d'une telle création dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial Nous nous étions abstenus sur le volet relatif à cette agence qui, dans l'attente de la remise du rapport Morvan, nous semblait prématuré. De même, nous avons rejeté l'amendement au projet de loi ÉLAN visant à créer cette agence par voie d'ordonnance. C'est pourquoi, après ces annonces présidentielle et gouvernementale qui promettaient un geste fort à l'endroit des territoires qui souffrent d'un manque d'ingénierie locale, nous sommes aujourd'hui surpris de constater que le Gouvernement n'a pas jugé utile de déposer lui-même un projet de loi, qui aurait été accompagné d'une étude d'impact et d'un avis obligatoire et public du Conseil d'État. C'est une proposition de loi émanant du groupe du RDSE qui nous est soumise, sur le temps réservé au Gouvernement, pour laquelle le Conseil national d'évaluation des normes, le CNEN, n'a pas été saisi. Les associations d'élus n'ont pas non plus été impliquées, ce qui révèle un manque de concertation très regrettable. Le Conseil d'État a rendu un avis, mais uniquement parce qu'il a été saisi de cette proposition de loi par notre président, Gérard Larcher. avis s'est d'ailleurs révélé très utile, car il a permis de corriger en dernière minute certains points techniques, dont la codification. La cohérence fait par conséquent défaut et la méthode employée nous laisse quelque peu perplexes quant à l'engagement du Gouvernement sur ce projet La création d'une agence de la cohésion des territoires répond donc à un véritable besoin exprimé par les élus locaux, afin de disposer d'un interlocuteur capable d'apporter des solutions opérationnelles à leurs problèmes, particulièrement dans les territoires fragiles, souvent les petites villes ou les milieux ruraux, qui manquent cruellement de ressources en termes d'ingénierie pour élaborer leurs projets. Les élus sont parfois découragés face aux difficultés qu'ils rencontrent parce qu'ils n'ont pas toujours les outils pour capter les appels à projets nationaux, pour dialoguer avec l'État et pour bénéficier pleinement des politiques publiques que celui-ci met en oeuvre. Tout cela n'est pas non plus facilité par la multiplicité de l'offre contractuelle qui leur est proposée : contrats de territoire, de ville, de ruralité, de revitalisation artisanale et commerciale, volet territorial des contrats de plan État-régions, contrats de site, de redynamisation, etc. La multiplication des interlocuteurs rend la coordination des actions complexe, d'où un besoin de clarification, de lisibilité et d'accompagnement par un État qui joue un rôle de facilitateur, permettant localement l'articulation de toutes les politiques publiques, quelle que soit leur origine. On trouve dans le rapport Morvan des préconisations particulièrement pertinentes à cet égard. Il recommande judicieusement un dispositif partant du projet de territoire, des besoins locaux et des demandes des élus, et s'appuyant sur des dispositifs d'État un contrat unique de cohésion territoriale, un dossier de financement unique, et la constitution d'équipes d'appui pluridisciplinaires. Ce rapport invite à une transformation nette de la relation entre l'État et les collectivités territoriales avec, dans le respect de la décentralisation, un État partenaire des collectivités pour faire aboutir des projets à l'échelon local.

Aucune analyse ne démontre la pertinence de la fusion d'opérateurs. Rien ne justifie que l'EPARECA et une partie de l'Agence du numérique se trouvent intégrés à l'agence par rapport aux autres opérateurs intervenant au profit des territoires. Notons de plus que l'exposé des motifs indique, et cela a de quoi susciter notre inquiétude, que le directeur général de l'agence devra présenter sous dix-huit un schéma de mutualisation des fonctions supports de tout ou partie des opérateurs mentionnés ». Un certain flou entoure le fonctionnement de l'agence. Nous aurons bien un interlocuteur unique en la personne du préfet dans le département, mais quelle sera la nature des relations contractuelles entre les territoires et l'agence ? Comment s'opérera l'articulation entre celle-ci, le préfet et les élus ? Comment l'agence se combinera-t-elle avec ce qui existe déjà et fonctionne bien dans certains territoires, comme les agences techniques départementales ? Enfin, et c'est une question essentielle, les prestations de l'agence seront-elles ou non facturées aux collectivités ? Nous avons aussi obtenu que, à terme, l'agence puisse disposer de fonds propres. Mais il n'est pas prévu de moyens supplémentaires autres que ceux des opérateurs qu'elle intègre et ceux qui proviennent de la Caisse des dépôts Elle fonctionnera à coût constant. Elle devra donc abandonner certaines missions existantes pour se consacrer aux nouvelles qui lui sont ainsi confiées. Nous proposerons donc, par nos amendements : de souligner le rôle de facilitateur que doit jouer l'État ; de positionner l'agence comme coordinatrice d'outils nationaux au service des territoires ; d'assurer qu'elle demeure une structure souple de garantir une gouvernance véritablement équilibrée ; de revoir la fusion des opérateurs ; de prévoir un dispositif renforcé au profit des territoires les plus en difficulté ; enfin, de s'assurer qu'elle puisse être saisie par toutes les collectivités. Je tiens aussi à relever la satisfaction du groupe socialiste sur deux avancées significatives votées en commission, que nous proposerons d'approfondir. La première concerne la gouvernance de l'agence. Une version proche de celle que nous avions proposée a été adoptée. Elle instaure un conseil d'administration composé de représentants de l'État et des collectivités territoriales en nombre égal, dans une logique de coconstruction donnant aux territoires toute leur place. Revenir sur cette parité entre l'État et les collectivités reviendrait à assumer une volonté recentralisatrice. Nous pensons au contraire que les collectivités doivent s'approprier l'agence et nous serons particulièrement vigilants sur cette question. La seconde consiste en la mise en place de comités de la cohésion territoriale au niveau départemental, réunissant les collectivités, leurs groupements, ainsi que les autres acteurs publics ou privés parties prenantes à la construction des projets de territoires. Ces comités auront pour objet de faire émerger des projets innovants et de suivre les projets soutenus par l'agence. Nous serons donc attentifs à leur maintien. Nous proposerons, pour compléter leurs missions, qu'ils ne se cantonnent pas au suivi de l'exécution des projets, mais qu'ils soient aussi informés des demandes émanant des collectivités. Pour conclure, mes chers collègues, nous nous réjouissons évidemment de la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires, qui répond à une véritable demande. Mais vous aurez compris que nous restons très réservés et interrogatifs quant au périmètre de cette agence, à son mode de fonctionnement et aux moyens effectifs dont elle pourra disposer. Nous craignons aussi la tendance recentralisatrice. Nous devons donc veiller à ce que l'agence ne puisse pas être au service du préfet dans une logique descendante, mais, bien au contraire, au service des collectivités dans une logique ascendante. Monsieur le ministre, avec Mme Gourault, vous avez pour mission de restaurer la confiance entre l'État et les territoires. Ne manquons donc pas l'occasion que présente cette proposition de loi pour y parvenir

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, animé par la volonté de représenter tous les territoires et de se faire le porte-voix des élus locaux, le groupe du RDSE a souhaité porter cette proposition de loi de création de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Vous le savez, face à la multiplicité des opérateurs, à la complexité des procédures et à la persistance de financements croisés, qui handicapent l'émergence des projets, les élus ont émis le souhait d'une meilleure lisibilité de l'ingénierie de projets. Nous sommes donc partis d'un double constat, celui du manque d'efficacité du système actuel et du besoin de mieux accompagner les territoires fragiles. Sur cette nous avons élaboré un texte permettant la création d'un guichet unique au service des élus locaux, afin d'accompagner les initiatives locales, c'est-à-dire rendre la décentralisation effective. Pour les collectivités ne disposant pas de l'ingénierie territoriale nécessaire, il s'agit d'un projet fondamental. Car ce sont bien les territoires les plus fragiles qui sont d'abord en attente d'une structure de conseil et de coordination. Ces dernières années, nombre d'entre eux n'ont pu faire émerger des projets par manque d'ingénierie et de moyens. Par exemple, les projets du dispositif Action coeur de ville, qui voient le jour partout en France, sont des opérations complexes et transversales pour lesquelles l'absence d'interlocuteur unique peut être un véritable frein dans certaines collectivités. Les élus locaux en sont bien conscients et sollicitent un choc de simplification. Cela a été rappelé, le Président de la République, lors de la première Conférence nationale des territoires en juillet 2017, puis devant le Congrès des maires, s'est dit « conscient de certains défis de la situation de déclassement des villes moyennes et de leur ruralité La création de l'agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, doit précisément répondre aux besoins des élus de terrain pour concrétiser, selon les mots du président Requier, « la promesse républicaine de l'égalité C'est dans cet esprit que notre groupe a souhaité porter cette proposition de loi. Je tiens ici à apporter quelques réponses aux inquiétudes qui ont émergé. D'une part, l'ANCT n'est pas en concurrence avec les agences d'ingénierie locales, elle leur est complémentaire, comme le permet aujourd'hui le droit de la concurrence. Elle n'a pas plus vocation à se substituer aux structures bien établies. Nous tenions à être parfaitement clairs sur ce sujet. Elle n'a pas non plus vocation à créer une charge supplémentaire pour les collectivités. Afin de l'inscrire dans la loi, le groupe du RDSE a déposé un amendement visant à préciser, à l'article 6, que les prestations de service susceptibles d'être facturées sont celles qui correspondent aujourd'hui aux missions industrielles et commerciales de l'EPARECA. D'autre part, grâce à la fusion du CGET, de l'EPARECA et de l'Agence du numérique, elle doit permettre à l'ingénierie locale d'être plus efficace, plus réactive, et d'en optimiser les coûts de fonctionnement. À moyens constants- le Gouvernement s'y est engagé -, l'objectif est de faire mieux et plus vite. Il s'agit bien de renforcer l'efficacité de l'intervention de l'État et de ses opérateurs, grâce à une meilleure coordination. En ce sens, nous avons déposé un amendement visant à supprimer la création des comités de la cohésion territoriale dans les départements, qui ajoutent de la complexité et nous apparaissent peu utiles et chronophages. Nous doutons par ailleurs du fait qu'ils puissent fonctionner sans aucuns frais et préférons assurer les élus d'une parfaite optimisation des financements. J'en viens ici aux deux points fondamentaux auxquels nous attachons une grande importance. S'agissant de la gouvernance de l'ANCT, nous sommes en accord avec le choix fait par la commission de donner plus de poids aux collectivités au sein du conseil d'administration. S'il s'agit bien d'une agence d'État, qui s'appuie donc naturellement sur le réseau préfectoral, elle doit avant tout son existence à l'initiative des collectivités et des élus. Nous proposerons d'ailleurs que l'outre-mer soit spécifiquement représenté. Cependant, nous nous étonnons de l'absence, au sein du conseil d'administration, de la Caisse des dépôts et consignations, qui joue pourtant un rôle essentiel dans le financement des projets. Nous vous proposerons donc de la réintégrer. J'en terminerai bien sûr par l'article 2, modifié en commission. Sur ce point, convaincus de l'importance du numérique sur nos territoires, nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale. Parmi les missions de l'Agence du numérique figure le plan France très haut débit, dont l'achèvement est prévu en 2022. Aussi, comme le Conseil d'État et le Gouvernement, nous croyons qu'il n'est pas opportun de reporter son intégration à 2021. Il faut au contraire inclure au plus vite l'Agence du numérique, dont les missions constituent une part essentielle du périmètre de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Reporter son intégration reviendrait à déstabiliser complètement l'édifice. Comment justifier cette absence, alors que la diffusion du très haut débit constitue aujourd'hui le coeur d'une grande partie des projets des territoires ? Quelle serait l'efficience d'une agence d'ingénierie dépourvue de prérogatives numériques ? Les risques sont élevés de voir l'ANCT devenir une coquille vide. Aussi, nous vous proposerons un amendement visant à fusionner dès 2020 le CGET, l'EPARECA et l'Agence du numérique. Monsieur le ministre, nous avons écouté Mme Gourault attentivement lors de son audition par la commission. Nous partageons l'ambition du Gouvernement de voir une agence pleinement opérationnelle dès 2020. Nous entendrons de nouveau avec grand intérêt votre désir de voir aboutir ce projet, tel qu'il est souhaité par les élus locaux, dans les plus brefs délais. Vous l'avez compris, le groupe du RDSE attend beaucoup des débats qui s'ouvrent, car c'est l'avenir de nos territoires, notamment les plus fragiles, qui est en jeu. Nous aborderons donc cette discussion avec la ferme volonté de faire de l'égalité des territoires une réalité. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'agence nationale de la cohésion des territoires va donc finir par voir le jour. Oubliant l'épisode imaginé par le Gouvernement de la création de cette agence un amendement au projet de loi ÉLAN en juillet dernier, les textes qui nous sont soumis aujourd'hui ont été déposés, avec l'aval du Gouvernement, par nos collègues du RDSE le 2 octobre dernier et font l'objet d'une procédure accélérée. Le Président de la République avait annoncé cette création devant l'ensemble des élus locaux le 17 juillet 2017 au Sénat à l'occasion de la première Conférence nationale des territoires, puis devant le Congrès des maires de France le 24 novembre 2017 alors qu'il annonçait la suppression progressive de la taxe d'habitation. Comme nous l'avait dit en commission la ministre Jacqueline Gourault, cette future agence était une demande de l'Association des maires de France, l'AMF, que le Gouvernement avait « écoutée Le président Macron précisait souhaiter que cette agence soit un « guichet unique » pour les collectivités, sur des sujets aussi divers que le numérique ou les déserts médicaux. De fait, l'aménagement du territoire ne peut être efficace que si l'on crée un pouvoir transversal, car nombre de sujets sont liés. Je relève au passage qu'il n'est plus question de faire de pont entre les ministères de la santé et de la cohésion des territoires, comme cela avait été évoqué à l'époque. Ce serait pourtant, à mon avis, la seule façon d'avancer vraiment sur le problème récurrent des déserts médicaux. La commission de l'aménagement du territoire du Sénat ne s'interdit toutefois pas de le traiter encore cette année à l'occasion de la discussion du projet de loi On note donc que, depuis juillet 2017, le processus de création de cette agence aura duré un peu plus longtemps que prévu. Il faut penser que l'opération n'était pas simple, malgré l'urgence à agir, dans un contexte de réduction sensible des dotations aux collectivités. Au-delà du sujet majeur des dotations qui a mis le feu aux poudres, il fallait évidemment entendre l'impatience des élus qui font, depuis de nombreuses années, partout remonter le fait qu'il y a trop d'interlocuteurs, trop d'opérateurs dans leurs démarches, trop de blocages, trop de délais. La vocation de l'agence est justement de « donner davantage de lisibilité et d'efficacité à l'intervention de l'État sur les territoires » par la voix des préfets qui en seront les « délégués territoriaux ». L'agence doit donc, « dans le respect du principe de déconcentration, contribuer à simplifier les relations entre les porteurs de projets locaux et l'État », en créant une structure dont la vocation serait d'accompagner les collectivités ayant de faibles moyens d'ingénierie et devant faire face à la grande complexité des procédures. Vaste programme, vous n'en doutez pas ! En clair, elle doit avant tout fluidifier les relations entre les élus locaux et l'exécutif et apaiser le dialogue au sein de la Conférence nationale des territoires. Une fois cela dit, beaucoup de questions restaient ouvertes et l'étaient encore dans les deux propositions de loi déposées. Je voudrais saluer à mon tour l'excellent travail de notre rapporteur Louis-Jean de Nicolaÿ pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : il a fait entendre la voix des élus locaux et proposé d'utiles enrichissements et rééquilibrages du texte, qui étaient nécessaires.

Les autres grands opérateurs- CEREMA, ANAH, ADEME et ANRU -ne seront pas intégrés dans l'agence, mais celle-ci sera appelée à « conventionner » avec eux. On le sait, car la ministre Jacqueline Gourault ne s'en était pas cachée lorsqu'elle avait été auditionnée par la commission, il s'agit notamment d'un problème social ce n'est pas la même chose d'intégrer dans la nouvelle agence de petites structures comme l'EPARECA ou l'Agence du numérique, qui ne comptent que quelques dizaines d'agents,

être l'occasion d'une rationalisation saine, une expression de la réforme de l'État dont on parle tant et dont on voit si peu de résultats. S'agissant des moyens et de la gouvernance, peu d'informations nous étaient données. Pour ce qui est de la gouvernance, il avait été dit initialement que « les élus locaux devraient jouer un rôle dans la gouvernance de l'agence mais que leur poids et leur mode de désignation allaient être négociés avec « les parlementaires et les associations d'élus et c'est heureux, sur l'initiative du rapporteur, nous avons sensiblement amendé le texte de l'article 3, en prévoyant que le nombre de représentants des collectivités devrait être égal à celui des représentants de l'État.

le rapporteur a fait part de nos craintes : « Le financement de l'agence ne saurait venir en soustraction de moyens actuellement accordés aux collectivités territoriales.

Comme le rapporteur, je souhaite que l'agence soutienne en priorité les projets innovants des collectivités territoriales, qu'il faut aider partout sur le territoire, en valorisant les beaux projets, que ce soit en matière de mobilités, d'alimentation saine, durable et de proximité, de reconquête de la biodiversité, de création de nouveaux espaces de vie commune. Pour conclure, reste à suivre évidemment les modalités d'installation de cet outil de décentralisation de la politique d'aménagement et de soutien aux territoires afin d'en concevoir l'utilité réelle. À cet égard, l'identité de son dirigeant, son parcours, son charisme et sa capacité d'entraînement seront fondamentaux. Il faudra que nous soyons très vigilants sur son profil.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de nombreux territoires se sentent délaissés, voire carrément abandonnés. Beaucoup de services se détériorent avant de disparaître progressivement des zones les plus isolées. Pourtant, les élus locaux se battent tous les jours pour préserver et développer leur territoire. Ils ne savent plus qui solliciter pour espérer obtenir une liaison téléphonique correcte, du très haut débit, ou des projets de réhabilitation ou de développement de plus grande ampleur. L'agence qui nous est proposée aujourd'hui vise à regrouper certains organismes et à assurer une meilleure coordination dans les projets.

Comment pourra-t-il faire face à cette charge nouvelle, sachant que les préfectures sont débordées et subissent déjà des réductions d'effectifs ? Est-il prévu que ces dernières disposent de moyens humains supplémentaires ? Sur quels organismes locaux le préfet pourra-t-il s'appuyer ? Bonne question ! Vous conviendrez que l'avancement des projets sera fortement lié à la personnalité et à la volonté propre de chaque préfet. Seront-ils tous en mesure de répondre à cette forte attente des territoires ? Par ailleurs, concrètement, nous aimerions savoir comment et dans quelles conditions l'agence proposera ses services. Conclura-t-elle des contrats avec les collectivités, avec comme intermédiaire le préfet ? Ses prestations seront-elles gratuites ? L'agence, donc le préfet, deviendra-t-elle un intermédiaire systématique entre les collectivités et les agences conventionnées ? Au contraire, sera-t-il toujours possible pour une commune ou un groupement de communes de saisir directement l'ANAH ou l'ANRU ? Si tel ? Si tel est le cas, à quoi servirait le conventionnement avec l'agence ? Nul doute que le débat qui va suivre permettra de répondre en partie à ces questions.

Enfin, il reste la question des financements de l'agence et des moyens alloués à ses actions. Il ne faudrait pas, par exemple, ôter la dotation d'équipement des territoires ruraux pour pouvoir bénéficier des services de celle-ci. Plus directement, nous espérons bien évidemment des financements nouveaux en faveur des territoires, et surtout des territoires ruraux. Ainsi, malgré toutes les interrogations qui demeurent, nous estimons que la création de l'agence doit être encouragée. Nous resterons vigilants sur l'application et la mise en place de ses actions. Monsieur le ministre, vous pourrez compter sur notre bonne volonté dans les territoires pour favoriser ces dernières. Pour conclure, vous le savez, les attentes des élus et des territoires sont très fortes. Nous espérons vivement que l'agence permette de répondre à certaines problématiques, concerne le très haut débit. Mais sachez que, si pour une raison ou pour une autre, l'action de l'agence se trouvait contrainte, notre déception en serait d'autant plus grande ! Très bien Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires a été évoquée à plusieurs reprises par l'Association des maires de France et par de nombreux groupes politiques. L'intention est bonne à condition que l'ensemble du processus soit parfaitement défini pour s'insérer dans une organisation durable de l'aménagement territorial. Il convient d'éviter une aggravation du phénomène du millefeuille institutionnel. Ce débat, au-delà de sa pertinence technique, révèle que les territoires attendent davantage d'attention des services de l'État. Il est évident que la République ne peut pas fonctionner sans une collaboration étroite entre l'État et les collectivités territoriales. La création d'une agence nationale de la cohésion des territoires doit permettre de lutter contre les multiples fractures- numérique, sociale, économique -qui traversent notre pays. Sur le principe, le groupe Les Indépendants - République et Territoires y est bien sûr favorable. Nous soutenons Nous soutenons tout ce qui peut renforcer notre cohésion nationale et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Toutefois, il faudra veiller à ce que ce nouvel acteur n'ajoute pas une couche de complexité bureaucratique au quotidien déjà bien encombré des élus locaux. Son périmètre large ne doit pas conduire à une dilution de son action, car qui trop embrasse mal étreint ! Les élus locaux attendent surtout de l'État une lisibilité globale et un accès facilité au profit de leurs territoires. La nouvelle agence doit impérativement porter cette ambition de simplification pour mieux répondre aux besoins et aider les élus de terrain. La réussite de l'agence dépend essentiellement de la représentation des élus locaux au sein de ses instances. Comment pourront-ils y participer ? Comment seront-ils désignés ? Les élus territoriaux doivent être le plus possible présents afin de contribuer directement aux choix stratégiques. Il est essentiel d'associer davantage les élus locaux à la gouvernance centrale de l'agence : nous soutenons l'instauration d'un comité local de la cohésion territoriale à l'échelle départementale. Si le préfet devient le correspondant unique des élus, quels seront les moyens complémentaires mis à sa disposition par l'agence pour organiser, sur le terrain, au quotidien, le soutien promis aux territoires ? Comment assurer l'accès à l'agence, la lisibilité et le contrôle de son action ? Enfin, cela Enfin, cela a été dit, l'agence doit se concentrer sur les territoires les plus en difficulté, incluant les zones de revitalisation rurale, de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Il convient que l'agence soit aussi déconcentrée que possible, au plus proche des élus et de leurs préoccupations quotidiennes. Ces thèmes nous tiennent à coeur et notre assemblée en a fait un axe majeur de son action législative ces derniers mois. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous nous suivrez sur cette voie. La mise en oeuvre d'une agence nationale de nombreuses interrogations. Rien ne serait pire qu'une nouvelle usine à gaz qui élargisse le fossé entre l'État et nos territoires. Nous devons proposer aux élus locaux que nous représentons une solution opérationnelle, pragmatique et surtout utile. La

La première, c'est que la France n'est pas un bloc de pierre monolithique qui pourrait être gouverné depuis Paris. Elle est faite d'équilibres et d'identités qu'il est important de respecter pour mieux créer son unité. La seconde, c'est que la non-prise en compte de la diversité des territoires et de leur avenir est l'un des enjeux majeurs de la crise française actuelle. J'en suis persuadé. Les enjeux de la cohésion des territoires, cette capacité à concilier la diversité des territoires et la réduction des inégalités entre citoyens liées à l'espace, sont donc fondamentaux. Nous devons nous mobiliser de manière conjointe- collectivités, élus locaux, État, et plus largement société civile -pour que la cohésion entre les territoires soit réelle et pour bâtir en commun un aménagement durable et innovant des territoires. est beau, mais quelle pourrait en être la traduction concrète ? L'agence nationale de la cohésion des territoires est un des éléments de réponse que nous étudions aujourd'hui, et je remercie le rapporteur Louis-Jean de Nicolaÿ, qui a travaillé sur ce texte. La présente proposition de loi se veut la concrétisation législative de la politique d'aménagement du territoire de l'exécutif. Pour reprendre les mots du Président de la République prononcés lors de la première Conférence nationale des territoires, la vocation de l'agence serait de fournir un « appui en particulier en ingénierie publique indispensable dans le rural et dans les territoires les plus périphériques » et de créer « une logique de guichet unique et de simplification de projets pour les territoires ruraux, les villes moyennes en difficulté

de plus de simplification. Mais la condition de la création de cette agence est qu'elle soit réellement au service des territoires, notamment des communes. J'insiste sur ce dernier point, monsieur le ministre : nous connaissons tous la situation des collectivités territoriales, et notamment des plus rurales, qui se sentent de plus en plus dépossédées

Ce texte présente certaines avancées : la création d'un guichet unique pour les collectivités territoriales, par exemple, est un souhait formulé depuis longtemps par les élus locaux. ce texte du Gouvernement ne répond pas aux espoirs soulevés par la mission de préfiguration voulue par le Premier ministre en personne. Même si la forme juridique de l'agence nationale de la cohésion des territoires ne pose pas de difficulté, des imprécisions subsistaient sur sa gouvernance et sur son format. la gouvernance, nous avons souhaité renforcer le poids des élus en créant un comité local de la cohésion territoriale et en instaurant, au sein du conseil d'administration, la parité entre représentants de l'État, d'une part, et représentants des élus locaux et nationaux, ainsi que des agents de l'établissement, d'autre part. La cohésion des territoires ne se fera pas sans les élus ni sans les parlementaires. Les élus connaissent parfaitement leur territoire. Ils doivent avoir toute leur place dans l'organisation de cette agence. J'ajoute que le lien entre parlementaires, élus locaux et État est indispensable pour le fonctionnement d'une démocratie représentative au service des territoires. Cette agence pourrait justement redonner des leviers d'action locale aux parlementaires. Depuis la suppression de la réserve parlementaire, qui était pourtant un outil indéniable pour créer de la proximité entre les parlementaires engagés sur des dossiers locaux et les maires et les conseils municipaux, le risque d'éloignement progressif entre les communes du territoire et le parlementaire est bien réel. nous avons souhaité garantir la prise en compte des territoires les plus fragiles en précisant les zones d'intervention de l'agence. De plus, pour assurer le succès de l'intégration de l'Agence du numérique à l'agence nationale de la cohésion cohésion des territoires, nous avons aménagé une période de transition en prévoyant son transfert au 1 janvier 2021. L'agence doit en effet constituer une réponse efficace, notamment en matière d'ingénierie, pour soutenir les territoires ruraux et périurbains traversés par des fractures-

ce qui a bloqué la vie locale. Dans ce type de situation d'urgence, les élus locaux veulent des interlocuteurs d'État prêts à agir immédiatement. véritable enjeu du numérique, c'est aussi de travailler à l'acculturation, aux ouvertures et aux potentialités pour attirer de nouvelles populations dans les départements et consolider l'économie actuelle.

Monsieur le ministre, les attentes des élus locaux et des citoyens sont grandes pour la cohésion de nos territoires. Nous devons à tout prix éviter la création d'une énième agence de type « coquille vide ». Nous appelons ainsi le Gouvernement à être particulièrement vigilant sur trois sujets : celui des ressources d'intervention dont bénéficiera l'agence, celui de la rationalisation des interventions de l'État dans les territoires

Mode de gouvernance néolibérale mis à l'honneur d'abord en. Grande-Bretagne, les agences, après les autorités administratives indépendantes- « États dans l'État », disait à l'époque Jacques Mézard -, sont à la mode.

L'IGF constatait alors que les dépenses et les effectifs de ces « agences » croissaient bien plus vite que ceux de l'État. Elle soulignait que « la constitution d'agences se traduit mécaniquement par une augmentation des coûts de structures des politiques publiques » le pilotage de l'État peut « conduire à bureaucratiser l'exercice de la tutelle ». Conclusion de l'IGF : la création des agences ne résulte pas d'une stratégie globale, mais de décisions prises au gré des opportunités, sans cohérence d'ensemble et sans analyse coûts-avantages de la gestion par agences plutôt que par l'administration classique. Toute ressemblance avec l'agence nationale de la cohésion des territoires ne serait pas totalement fortuite ... Il faut répondre au mécontentement des élus, paralysés par des réformes stupides, et, en même temps, faire des économies et libéraliser ? Faisons donc une agence et célébrons à son de trompe trompe cette colossale innovation, plutôt que de donner à l'administration territoriale les moyens de ses missions. Si cette bonne idée donne les mêmes résultats que les réformes adoptées depuis 2010, mes chers collègues, nous avons du souci à nous faire

le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Toutefois, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, ruraux ou urbains.

Dans ces conditions, et parce que les ambitions de la cohésion des territoires sont rappelées régulièrement par le Gouvernement, l'agence nationale de la cohésion des territoires a vocation à s'installer dans une ville moyenne.

quel plus beau symbole que d'installer cette agence au service de l'ensemble des territoires de notre pays là où le Gouvernement a réaffirmé, le 14 décembre 2017, la prise en compte par l'État de cet enjeu territorial majeur pour la France, c'est-à-dire à Cahors Édouard Philippe s'était alors enorgueilli de mettre en place une nouvelle « grammaire » des relations entre l'État et les collectivités territoriales dans la ville natale de Clément Marot, créateur, au XVI siècle, de la fameuse règle de l'accord du participe passé. La parole

de l'ingénierie confrontée à des modèles de développement et au savoir-faire citoyen. Les développeurs d'hier et d'aujourd'hui n'ont plus le monopole, tant s'en faut, du développement territorial. Il faut entendre et voir la diversité de ceux qui y contribuent. Il n'y a pas de monopole de l'ingénierie. Deux conceptions peuvent en effet se confronter et doivent s'organiser : d'un côté, l'aménagement pour les territoires- vision plus technique et descendante de l'ingénierie des territoires qui nous réunit aujourd'hui de l'autre, l'aménagement par les acteurs- vision collaborative portée et accompagnée par une ingénierie territoriale d'animation. Le développement local, notamment en territoire rural, s'est souvent lancé le défi de concilier ces approches dans une démarche collaborative au service de la construction du projet intégré de territoire local. L'usage, l'expérience, la connaissance par chacun de la réalité locale trouvent ici toute leur place. L'ingénierie a muté. Il ne s'agit plus d'accompagner, voire de porter des projets, mais de faciliter la rencontre, la médiation et même l'intermédiation entre des élus qui se professionnalisent, des entreprises qui se mondialisent ou se territorialisent et des citoyens et acteurs sociaux de plus en plus en demande de participation et d'investissement social local. ingénierie solide est donc avant tout collaborative, coopérative, associant une diversité d'acteurs, d'élus, de citoyens, de professionnels pour faire émerger des projets territoriaux robustes adaptés au potentiel des entités locales et articulés avec les territoires voisins. Il ne s'agit donc pas, à travers la mise en place d'une agence- et j'appelle à la vigilance sur ce point -de bureaucratiser l'ingénierie territoriale, mais, bien au contraire, de l'organiser selon une approche décentralisée et partenariale. La

Je sens bien que l'État, à travers cette agence, essaie de renouer le dialogue avec le territoire.

de composer avec le phénomène de métropolisation au bénéfice des territoires hors métropole, nous n'arriverons à rien ! On pourra créer toutes les agences que l'on veut,

aux collectivités territoriales dites « infra », à savoir les syndicats, les EPCI et les communes. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai signé une circulaire destinée à l'ensemble des préfets de France, qui doivent faire remonter tous les « irritants » liés à l'application de la loi NOTRe. La situation pose d'ailleurs très clairement la question